L'ordre du jour appelle la nomination des 27 membres de la mission d'information sur le thème : « Enjeux de la filière sidérurgique dans la France du XXI siècle : opportunité de croissance et de développement », créée sur l'initiative du groupe Union Centriste en application du droit de tirage prévu par l'article 6 du règlement.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

Nous venons d'avoir ce débat en commission spéciale voilà quelques minutes, et je souhaite le prolonger dans l'hémicycle. Depuis hier,

En réponse à votre rappel au règlement, monsieur Gay, et pour éclairer tous nos collègues, je souhaite préciser que l'article 48 du règlement du Sénat confie à la commission saisie au fond d'un texte la mission de se prononcer sur la recevabilité des amendements au titre de l'article 45 de la Constitution. Sont seuls recevables les amendements qui s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent ou, en première lecture, ceux qui présentent un lien, même indirect, avec le texte en discussion. Ce contrôle de recevabilité qui nous incombe concerne autant les amendements des sénateurs que ceux du Gouvernement.

par rapport au texte issu des travaux de l'Assemblée nationale ou par rapport à l'intitulé d'un texte. Pour cette raison, sur l'initiative des rapporteurs, la commission a d'ailleurs supprimé des articles nouveaux introduits dans le projet de loi par nos collègues députés.

-, la fiscalité des entreprises- sauf si la disposition se rattache à un sujet du texte initial, comme la fiscalité sur les jeux -, les règles de la commande publique, le droit du travail-

M. Gay a lui-même évoqué ce problème lors de la discussion générale en disant à juste titre que ce texte contenait dix projets de loi à lui tout seul ! Évidemment, ces déclarations d'irrecevabilité ne préjugent pas l'appréciation que l'on peut porter sur le fond des amendements concernés.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, comme je m'y étais engagée en commission, j'ai travaillé à une rédaction qui préserve les emplois menacés en France, mais qui soit également conforme à la future directive européenne. Je rappelle que ce projet de loi entend lever les freins à la croissance des entreprises. Il s'agit en l'occurrence de libérer les entreprises françaises du secteur de la plasturgie de contraintes qui ne s'appliqueront pas à leurs concurrentes européennes.

qui sont bien appliquées par les industriels, et revient uniquement sur les dispositions les plus excessives et les plus floues de la loi ÉGALIM, tout en transposant très exactement la nouvelle directive en passe d'être définitivement Je vous propose également de limiter l'interdiction des contenants en plastique dans les cantines, issue de la loi ÉGALIM, aux seuls usages de cuisson et de réchauffe. Le

aux difficultés industrielles qu'entraîne, en particulier, l'interdiction des couverts en plastique à très brève échéance. Je connais bien le cas de cette entreprise du Loiret dont nous a parlé M. Cardoux. Malgré ma réserve sur la compatibilité avec le droit européen, je m'en remettrai donc à titre personnel à la sagesse du Sénat sur le sous-amendement n° 944 rectifié, qui prévoit une exception limitée dans le temps pour les couverts compostables et constitués

! Au moment où une grande réforme de la Constitution se prépare et où le droit d'amendement pourrait être mis à mal, on ne peut pas à

En effet, nous évoquions à l'époque la problématique des sacs plastiques à usage unique et des films de routage. Nous évoquons aujourd'hui les gobelets, les pailles, etc. Mes chers collègues, je pense très sincèrement que nous devrions arrêter ce que nous pourrions appeler le « plastique ». Je suis élu d'un département, la Haute-Loire, où le secteur de la plasturgie génère plus de 2 000 emplois. Dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes, chère à Mme la rapporteur, plus de 500 entreprises interviennent dans ce secteur d'activité. Ce sont des Ce sont des industriels qui ne cessent de faire évoluer leurs process grâce à la recherche et au développement, notamment sur les matières biosourcées, largement évoquées. Ce sont des industriels qui sont conscients des enjeux environnementaux et qui développent des filières de valorisation et de recyclage. Ce sont aussi des entreprises qui recrutent des opérateurs, mais également des techniciens de très haut niveau. Alors, de grâce, madame la secrétaire d'État, à la veille d'une énième directive européenne, laissons le temps à cette activité de pointe de s'adapter.

la Haute-Loire. Il faudra un certain temps pour que les industriels qui ont toujours travaillé le plastique à base de pétrole travaillent le plastique à base de produits biosourcés. Mais on va dans

Merci

Dès lors qu'un texte évoque la croissance et la transformation des entreprises, il ne me paraît pas anormal qu'une majorité de sénateurs qui mettent en doute

mais dans cette affaire, j'ai plus d'interrogations que de certitudes. Je demande le droit au doute, non pas sur ce sous-amendement, mais sur la manière dont nous abordons le problème.

Comment imaginer que des entreprises, qui ont investi pendant des années dans des process extrêmement lourds, vont pouvoir en deux ou trois ans transformer complètement leur production ? Cela n'est pas possible. Il faut leur donner du temps, comme l'ont dit certains. Je vous

Cet amendement s'inscrit dans la suite de la discussion que nous venons d'avoir, même si le sujet est différent. Je ne suis pas de ceux qui souhaitent voir la transition écologique retardée, mais je pense, comme d'autres dans cet hémicycle, qu'il faut procéder avec méthode et organiser cette transition en tenant compte de son incidence sur les territoires

qui ne sont plus autorisés en Europe, mais qui sont commercialisés en dehors de celle-ci. La directive européenne qui régule ce secteur n'a pas décidé de revenir sur cette commercialisation à l'extérieur de l'Union européenne.

que les pays qui utilisent ces produits n'hésiteront pas, en cas d'interdiction de la commercialisation en France, à aller les acheter chez nos voisins allemands, italiens et espagnols, qui continueront de les produire. J'ajoute que la transition est secteur. Il faut l'accompagner. Ces entreprises, notamment les plus importantes, se sont engagées dans la diversification de leurs productions et prévoient des investissements massifs dans l'agro-écologie, en particulier dans les techniques de biocontrôle. Nous devons leur laisser le temps de s'organiser en transformant les emplois pour les pérenniser.

J'ajoute que l'interdiction ainsi opposée aux fabricants français sera strictement sans effet sur l'utilisation de ces produits dans les pays tiers, lesquels

Gouvernement ? Ces amendements identiques visent à abroger l'interdiction de fabrication sur le territoire français de produits pharmaceutiques, dont l'usage n'est pas permis au sein de l'Union européenne, et destinés à être commercialisés dans des pays situés hors de l'Union, où leur utilisation est autorisée.

auprès d'autres producteurs au sein de l'Union européenne ou dans des pays tiers, ce qui conduit à s'interroger sur cette mesure et son objet. Vous le savez, le Gouvernement soutient l'objectif de réduction dans le monde de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques interdits à la consommation au sein de l'Union européenne. La question soulevée par le Sénat concernant l'emploi industriel- plus de 1 000 emplois directs et, potentiellement, jusqu'à 3 000 emplois au total -est néanmoins importante, et n'avait pas fait l'objet d'une étude d'impact lors de l'adoption de cette mesure à l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi ÉGALIM. Dès lors, la discussion doit pouvoir se poursuivre sur cette mesure, afin d'en adapter la

N'oublions quand même pas que près de 80 % de l'alimentation mondiale est produite par la petite agriculture familiale, qui n'utilise pas du tout de produits chimiques. Cette agriculture mérite d'être accompagnée

question de respect des textes que nous avons votés. Avec la loi sur la biodiversité, nous avons inscrit dans le code de l'environnement le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement

du Sénat. J'espère que notre assemblée sera à la hauteur de sa réputation. La parole

que l'on peut les acquérir auprès de l'Espagne, de l'Italie et de l'Allemagne, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis pour l'Europe, à condition que ce soit toute l'Europe et que les règles s'appliquent à tout le monde dans les mêmes termes. La

Pour la majorité des salariés, on considère que tout travail entre 21 heures et 7 heures du matin constitue du travail de nuit. Le code précité a prévu une exception pour certaines catégories de métiers, l'intervalle est restreint, le travail de nuit n'étant pris en compte qu'entre minuit et 5 heures du matin. Cette exception est justifiée par la nécessité, pour certaines professions, de maintenir leur activité pendant la nuit. C'est le cas pour la presse, la radio, la télévision, le spectacle vivant, les discothèques, etc.

Ces règles sont souvent perçues comme des contraintes et des coûts supplémentaires pour les entreprises, alors qu'elles ont un but bien précis : protéger les salariés en leur assurant un droit au repos et en préservant leur santé et leur sécurité. Pourtant, depuis plusieurs années, les mesures de dérégulation du travail se multiplient. Après la loi Rebsamen, la loi Macron, la loi El Khomri et les ordonnances du 22 septembre 2017,

introduites dans un prochain projet de loi.

Il n'y a pas de raison de s'aligner sur les Galeries Lafayette et le Printemps

qu'après délibération du conseil municipal. J'ai interrogé plusieurs ministres sur ce sujet, m'étonnant de la sollicitation de la compétence d'un maire sur un accord partenarial : il en est ainsi.

de soutenir les centres-villes et les centres-bourgs en permettant de limiter ou, en tout cas, de gérer à l'échelon local

vingt ans, de définir le nombre de dimanches et de jours fériés où les grandes surfaces alimentaires périphériques sont ouvertes. Cela, naturellement, ne concerne pas les zones d'activité touristique. Je pense donc, madame la secrétaire d'État, que la vertu que le Gouvernement prône sur ce sujet, la cohérence et l'actualité

et à leurs élus la responsabilité d'apprécier l'opportunité d'ouvrir ou de fermer des grandes surfaces qui font évidemment de l'ombre à nos petits commerces. Si elles restent ouvertes quand nos petits commerces le sont aussi, il va de soi que la clientèle se précipitera davantage vers ces grandes surfaces, dans lesquelles ils vont déjà toute la semaine.

on ne peut qu'être solidaire de l'engagement de ces élus locaux et des finances locales. Or on les met en péril, dès lors qu'on les confronte à la puissance de feu des grandes surfaces,

prévoit que « le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés et après avoir recueilli, dans le secret de l'anonymat, la volonté de la majorité des membres de la profession, ordonner la fermeture au public ». Une large concertation est donc prévue, qui respecte parfaitement les textes qui régissent le commerce dans notre pays.

madame, monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, plusieurs articles de ce projet de loi suppriment des sur-transpositions de directives européennes.

visant à revenir sur les sur-transpositions réglementaires pesant sur la compétitivité des entreprises françaises. Le 7 novembre dernier, le Sénat a adopté le modeste projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français,

Il est souhaitable que, dans le cadre du projet de loi PACTE, nous n'ayons pas à écouter trop de chants de sirènes corporatistes ! L'article 9 de ce projet de loi aligne l'obligation de certification des comptes sur les seuils européens, seuils bien plus élevés que les nôtres. Avec les seuils européens, seulement 46 000 entreprises allemandes ont l'obligation de recourir à un commissaire aux comptes, contre 182 500 en France. Or tous ceux qui connaissent l'économie allemande savent que les entreprises sans commissaires aux comptes ne sont pas source d'une insécurité juridique, fiscale et commerciale particulière. Avec sagesse, la commission spéciale a tenu bon, en dépit des interventions des commissaires aux comptes. Nos PME, qui croulent sous les charges, pourront ainsi faire l'économie d'une dépense estimée en moyenne à 5 500 euros. Avec le projet de loi PACTE, nous avons l'occasion de mettre nos actes en conformité avec nos discours dominicaux

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le moins que l'on puisse dire de cet article, ouvrant le chapitre du projet de loi relatif à la réforme du commissariat aux comptes et de la profession d'expertise comptable, c'est qu'il va faire débat Il faut dire que cette réforme a déjà été testée dans un certain nombre de pays européens, fort divers quant à leur histoire administrative et fiscale- Portugal, Suède, Italie -, et que les premières évaluations n'ont pas été tout à fait probantes. Que la réforme de l'expertise comptable provoque quelques hésitations dans un pays comme l'Italie, où l'appareil statistique existant est parfois défaillant pour déterminer la réalité de la production économique et, partant, l'exacte contribution du pays au budget européen et à quelques institutions communautaires bien connues, devrait presque suffire, mes chers collègues, à nous alerter quant aux risques que nous encourons à transposer ces directives européennes

Les entreprises dont l'effectif salarié dépasse le seuil de 50 salariés, celui constituant l'un des critères de la réforme, se comptent en un nombre plutôt réduit : 35 000. La zone d'ombre, si l'on peut dire, ce sont les entreprises dont l'effectif salarié se situe entre 10 et 49 salariés, pour lesquelles il est probable que le critère de chiffre d'affaires ou de bilan puisse justifier de les faire entrer dans la catégorie des entreprises dispensées.

N'oublions pas que les trois quarts de nos entreprises sont des prestataires de services sans production industrielle. Nous sommes donc plus que réticents à l'adoption de cet article. La parole l'un des principaux arguments retenus par le Gouvernement pour aligner la France sur les seuils européens en matière de nomination de commissaires aux comptes est la création d'emplois. Quand on sait que les honoraires moyens d'un commissaire aux comptes dans une PME sont de 5 000 euros, soit 3 500 euros après déduction de l'impôt sur les sociétés, on se demande,

un commissaire aux comptes qui décèle une tentative ou une volonté de fraude fiscale ou d'évasion fiscale dans une entreprise sait faire preuve de persuasion et, croyez-moi, la crainte du commissaire aux comptes joue parfaitement. Par conséquent, on ne peut pas quantifier les « économies » de fraude fiscale que l'on réalise ainsi.

Résultat, ces sociétés se tourneront vers les grands cabinets, les anciens ou les autres, qui, une nouvelle fois, trusteront les mandats de commissaire aux comptes. Aussi, ce centre d'activités se situera dans les métropoles et ne créera plus d'activités en milieu rural.

qui prévoit de relever les seuils de certification légale des comptes par un commissaire aux comptes. Cette disposition menace sérieusement la sécurité financière des petites et moyennes entreprises, qui ne seront plus incluses dans le giron de la certification.

ne semble pas apporter de valeur ajoutée suffisante au droit français en matière de publicité des comptes sociaux de nos entreprises et ne doit donc pas être retenu. Il serait dommage que, pour rejeter une supposée sur-transposition, nous nous retrouvions avec une fenêtre supplémentaire de fraude et d'évasion fiscales.

Qui peut nous faire croire qu'une entreprise qui réalise 3 millions d'euros de chiffre d'affaires ne peut pas supporter 3 500 euros d'honoraires ? Qui peut nous faire croire qu'il faudrait faire plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires pour supporter 3 500 euros d'honoraires ? Qui a donc inspiré cette mesure ?

madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs,

eu lieu. De manière plus générale, je comprends que l'on s'inquiète d'une insuffisante étude d'impact. Peut-être tous les documents ne vous sont-ils pas parvenus, mais c'est l'un des articles pour lequel le dossier est le plus étayé et le plus complet. Comme vous le savez, cette réforme s'inscrit dans une vision globale : elle part d'une mission de l'Inspection générale des finances, qui a examiné le bien-fondé de ces seuils, puisqu'il s'agit d'une sur-transposition, sujet

3 500 euros pour une entreprise sous les seuils européens, et pèse plus lourdement pour les petites entreprises, rapporté à leur chiffre d'affaires et, surtout, à leurs résultats, donc à l'argent qu'elles gagnent effectivement.

Enfin, l'obligation d'audit légal pour les entreprises sous le seuil européen n'améliore pas l'accès des entreprises aux financements. La suppression de l'obligation de faire auditer les comptes signifie une économie de près de 700 millions d'euros pour les PME. Ce n'est pas rien

et l'expérience montre- je peux le confirmer par mon expérience personnelle, puisque nous avons tous des expériences antérieures -que, sur des petites entreprises ou des petites unités, le travail de l'expert-comptable et celui du commissaire aux comptes C'est bien cela qui est visé. En revanche- et c'est tout le travail de concertation avec la profession des experts-comptables et des commissaires aux comptes -, nous avons formulé des propositions pour rééquilibrer cette mesure de façon à à ce que les commissaires aux comptes puissent travailler sur des missions à valeur ajoutée pour les entreprises, la mission d'audit simplifié pour les petites entreprises, la mission d'audit pour les petits groupes. Je n'entre pas dans les détails, vous connaissez tous ces éléments : ils sont dans le texte équilibré que nous vous

Nous sommes dans une situation étonnante. Nous avons discuté pendant près de deux heures sur un certain nombre d'amendements en condamnant les sur-transpositions

et le chiffre d'affaires, le Sénat s'érige en défenseur de la sur-transposition des seuils pour les commissaires aux comptes.

en est bien conscient- les commissaires aux comptes eux-mêmes, même s'ils n'ont pas peut-être pas été les premiers à le dire, l'ont reconnu -, cette profession n'a pas évolué comme elle aurait dû le faire ; elle n'a pas suivi l'évolution de l'économie et elle ne rend pas les services qu'elle devrait rendre aux entreprises.

reprenant d'ailleurs, comme cela a été dit à plusieurs reprises, une fonction d'expert-comptable, qui existe déjà, et rende d'autres services

avoir assisté à un certain nombre de débats avec des représentants des différents mouvements des commissaires aux comptes, je crois aujourd'hui entrés dans le processus de réforme de la profession. Un certain nombre d'engagements ont été pris par le Gouvernement

Le commissaire aux comptes a une mission légale, qui est définie par le législateur. S'il considère que les comptes ne sont pas sincères et véritables, il ne les certifiera pas ; il formulera

Merci rapidement sur des points qui ont été débattus, notamment sur les propos de notre collègue Henno. Cela ne fait pas de doute, la réforme telle qu'on l'envisage donnera la main aux cabinets anglo-saxons.

d'une manière très fidèle toutes les observations formulées par les petits cabinets de province. C'est un dilemme qui existe depuis des années, les compagnies nationales sont à la main des cabinets anglo-saxons : je l'ai subi, je l'ai pratiqué et je peux l'affirmer. Quelle est la différence entre ces deux approches

J'arrive le lundi matin au cabinet, j'ai un casier, je l'ouvre, je trouve une enveloppe, je ne sais pas où je vais, il y a un billet de train, le nom de la société et j'y vais, je ne connais pas les dirigeants, je ne connais personne, je vais faire de l'audit intégral. » Est-ce cela la relation de proximité que l'on veut entre les professionnels du chiffre les entreprises ? Là, on va avoir une approche tout à fait anglo-saxonne, au détriment du lien humain et du lien de proximité, et on va une fois de plus dépouiller les territoires.

-, aussi bien celui de la compagnie locale des commissaires aux comptes que celui de l'ordre des experts-comptables : cette mesure fera fondre de manière extrêmement sensible l'activité des cabinets, et ce n'est pas une question de rente. On va me dire qu'ils sont assis sur des rentes ... Mais moi je parle de rente de survie dans les territoires dont je viens de donner les indicateurs majeurs.

les jeunes dont on a encouragé la formation, car, il y a quelques années, le métier d'expert-comptable et celui de commissaire aux comptes étaient des métiers en tension : il n'y avait pas de collaborateur disponible. Des filières très professionnelles se sont ouvertes, sont ouvertes, et des jeunes peuvent aujourd'hui être des comptables et des commissaires aux comptes de haut niveau, grâce à cette incitation et aux efforts qui ont été fournis aussi bien par l'État que par les collectivités locales pour encourager ces formations.

des personnes qui travaillent et pour qui, souvent, traverser la rue pour trouver un emploi revient à tomber à la mer.

d'affaires, niveau que certains pays voisins n'ont pas voulu retenir au moment de la transposition de la directive de 2003 et ce, alors même que, dans d'autres domaines, les contrôles sont autrement plus sévères. Ainsi demande-t-on tous les trois mois à tout chômeur inscrit sur les listes de Pôle emploi ou à tout allocataire du revenu de solidarité active d'apporter la preuve des efforts

En 2015, la productivité moyenne par salarié était de 300 000 euros environ en termes de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 6 millions d'euros pour une entreprise de vingt salariés.

Mon amendement vise à exclure les entreprises des départements et régions d'outre-mer du dispositif de relèvement des seuils pour la nomination d'un commissaire aux comptes. En effet, compte tenu de l'étroitesse de ces territoires, le nombre d'entreprises répondant aux critères de l'audit légal est réduit. Le relèvement des seuils aurait pour effet de supprimer environ deux tiers des mandats actuels, mettant en péril l'activité des commissaires aux comptes dans ces collectivités, et engendrant une diminution du nombre de professionnels, ce qui pourrait se révéler nuisible pour la qualité du service rendu aux entreprises qui demeureront soumises à un audit de leurs comptes.

dont bénéficient les entreprises ultramarines, notamment pour leurs investissements productifs, justifient également le maintien des seuils actuels

Cette mesure est de nature à alléger les contraintes pesant sur les entreprises et à les aligner sur les exigences minimales du droit européen. Toutefois, elle fait encourir deux risques. Le premier concerne la pérennité des entreprises. La France possède deux fois plus de PME ayant entre 3 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires que l'Allemagne. que l'Allemagne. Les PME dans notre pays ont en effet une taille plus modeste. En exonérant totalement ces sociétés d'audit légal, nous risquons de laisser un nombre considérable d'entreprises sans regard extérieur et de favoriser ainsi un laisser-aller comptable, qui mettrait en péril la santé financière de ces sociétés et, par conséquent, l'emploi de leurs salariés. Le second risque concerne les finances publiques. Une PME dont le chiffre d'affaires est de 3 millions d'euros rapporte 600 000 euros de TVA. La perte de recettes fiscales que cette absence d'audit légal pourrait engendrer serait par conséquent considérable. Pour y remédier, les auteurs de l'amendement proposent de soumettre les entreprises réalisant moins de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires à un audit légal simplifié, dont le tarif serait plafonné à 2 000 euros hors taxes pour celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 et 5 millions d'euros,

dont l'objectif est précisément de protéger les salariés et de leur donner accès à une information de qualité sur les données comptables de l'entreprise. Ce point me semble donc déjà couvert par la législation en

correspondre à une mesure de protection de ces actionnaires minoritaires. Qu'est-ce qu'un actionnaire minoritaire dans une PME ? Dans le cas d'un groupe familial prêt à éclater, demander la certification des comptes, c'est déjà rassurer sur la valeur de la société ou sur son résultat.

M. Richard Yung. Cet amendement vise à permettre, aux sociétés anonymes qui ne sont pas soumises à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes, d'en désigner un spécifiquement

pour présenter l'amendement n° 481 rectifié. Le relèvement des seuils pour désigner un commissaire aux comptes risque de laisser les groupes de sociétés à filiales nombreuses sans contrôle légal des comptes, à l'exception de ceux de la société mère. Ce n'est pas un cas d'école : je pense, par exemple, aux groupes hôteliers ou aux groupes d'établissements de santé. En effet, l'alinéa 32 de l'article 9 du projet de loi prévoit la nomination d'un commissaire aux comptes dans les seules filiales représentant une proportion, fixée par décret en Conseil d'État,

amendement vise à mieux sécuriser les groupes de sociétés à filiales multiples, en imposant le contrôle légal d'un commissaire aux comptes dans leurs filiales, par ordre décroissant, jusqu'à atteindre 70 % du chiffre d'affaires agrégé du groupe. Pour faciliter l'évaluation de ce périmètre d'audit, il est proposé d'atteindre les 70 % de couverture en contrôlant en priorité les filiales les plus contributives, par ordre décroissant. Cette

le projet de loi PACTE risque de faire disparaître du périmètre de contrôle par un commissaire aux comptes bon nombre de filiales de groupes français, mais aussi et surtout étrangers. Un amendement, approuvé par nos collègues députés, a tenté d'introduire un seuil de chiffre d'affaires de la société contrôlée à 50 % du chiffre d'affaires du groupe pour déclencher l'obligation d'audit. Ce seuil sera totalement inefficace pour les groupes composés de multiples filiales. La commission spéciale du Sénat a essayé de corriger cette problématique, en introduisant un nouveau seuil : si la société contrôlée dépasse une proportion, fixée par décret, du chiffre d'affaires, du total du bilan ou de l'effectif du groupe. Ce nouveau seuil risque d'être tout aussi inefficace pour les groupes composés d'une multitude de petites filiales.

avec une logique pratique de taux de couverture sur l'ensemble des sociétés d'un même groupe, la rédaction proposée s'avère difficilement opérationnelle. La raison en est simple : ces amendements s'appuient sur la mention, juridiquement inconnue, de sociétés contrôlées les plus contributives,

rien ne justifie qu'un décret fixant un simple seuil et ne soulevant aucune question juridique spécifique soit soumis à un avis du Conseil d'État, qui rallongera d'autant le délai d'adoption du texte. Nous sommes également favorables

n° 249 rectifié. L'obligation de désigner un commissaire aux comptes dans les filiales de petits groupes a déjà fait l'objet de longs débats à l'Assemblée nationale, débats au cours desquels il est apparu qu'une telle obligation était utile. Elle permettrait d'introduire un regard extérieur sur les filières les plus importantes de petits groupes, dont la structure peut être complexe.

Cette mesure semble être du plus parfait bon sens, ne serait-ce que pour la protection des intérêts de ces actionnaires. Oui, madame la secrétaire d'État, nous sommes aussi attentifs à la destinée des actionnaires, non par démagogie, mais tout simplement parce que leur nombre pourrait très bien s'élever dans les années à venir, notamment si les salariés, au travers de l'intéressement et de la participation, deviennent les actionnaires obligés de leur propre employeur. Pour en revenir au sujet, vous conviendrez qu'il serait tout de même assez complexe, pour ne pas dire plus, qu'une entreprise de 20 ou 30 salariés mette en place un dispositif d'actionnariat salarié, d'épargne salariale ou encore d'épargne retraite sans déposer de comptes certifiés.

Comme le disait voilà peu un commissaire aux comptes, on va essayer de « limiter la casse » ! Nous l'avons vu, quelques emplois directs dans la profession du chiffre sont remis en cause avec cette réforme, qui risque, notamment, de ruiner les cabinets intervenant dans les bassins d'emploi privés de locomotive industrielle et employant plusieurs centaines de salariés. Ici, il s'agit de permettre aux salariés, dès lors que leur entreprise compte au moins 11 personnes employées, de demander- par exemple par la voix de leur délégué du personnel, quand il existe -la nomination d'un commissaire aux comptes pour leur entreprise. Au moment où d'aucuns s'interrogent sur l'éthique de l'entreprise et sa place dans la société, autant donner ce droit, relativement simple d'application, aux salariés Outre ces considérations, il est évident que les entreprises ont tout intérêt à pratiquer le jeu de la transparence, y compris avec leur propre personnel. Si tel est le cas, toute stratégie de changement pourra s'appuyer sur des données fiables et admises par toutes et tous. Le commissariat aux comptes, fidèle reflet de la situation,

qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ». L'alinéa 27 de l'article 9 vise donc à dispenser les commissaires aux comptes de produire la moindre observation sur les comptes de l'entreprise certifiée et, plus encore, à encourager les entreprises à s'en passer. Une telle démarche prive de fait les entreprises d'un avis extérieur,

cette analyse ne peut procéder que d'un travail mené indépendamment d'un engagement dans son actionnariat. On notera également que la question de confiance est posée auprès des tiers, dès lors que l'information peut manquer sur les capacités de telle ou telle entité à faire face aux défis du temps. Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que rejeter les termes

Sous couvert d'assurer une meilleure défense des intérêts économiques des entreprises françaises, l'article L.232-25 du code de commerce a organisé les conditions d'un véritable recul social-

de l'amendement n° 610, hormis le fait que cette question est traitée à l'article 13 du projet de loi, sur le fond, la confidentialité est bien entendu utile à l'égard des concurrents et je rappelle que le dépôt du compte de résultat demeure obligatoire. L'avis est défavorable.

De la même manière que le droit commercial laisse aux PME la faculté de publier ou non leurs comptes sociaux, il convient de leur laisser le droit de déterminer si elles ont besoin du concours d'un commissaire aux comptes. Le rapport du comité d'experts présidé par Patrick de Cambourg nous en donne les raisons. « En tenant compte du relèvement des seuils de désignation des commissaires aux comptes au niveau européen, [on constate] que ne seront plus soumises à la certification légale des comptes environ 24 000 SA sur les 32 000 recensées par l'INSEE en 2016, soit 75 % des SA qui y étaient soumises, et environ 25 000 autres sociétés commerciales- SARL, SAS, SNC, soit 20 % de celles qui y étaient jusque-là soumises. « Ce sont autant entreprises qui ne bénéficieront plus de l'alerte du commissaire aux comptes. « D'autres éléments peuvent être pris en compte pour parfaire l'estimation : actuellement un millier d'entreprises en procédure collective ont un effectif compris entre 20 et 50 salariés et/ou réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 3 millions d'euros. Si on exclut les SARL de cette dimension, ce sont 650 à 700 entreprises qui sont potentiellement concernées. À ces entreprises, pourraient s'ajouter plus de 400 défaillances supplémentaires- soit environ 60 % de plus. En conclusion, si en termes absolus le nombre des entreprises concernées peut paraître faible, en termes économiques, celles-ci représentent potentiellement 10 000 emplois menacés, ce qui correspond à 6 % du total des emplois menacés en France en 2017. Une telle situation constitue à l'évidence un sujet de préoccupation. Les magistrats que le Comité a auditionnés ont été unanimes pour déplorer cet impact du relèvement des seuils. « La question de l'alerte est délicate pour les entreprises qui ne sont pas ou ne seront plus soumises à la certification légale obligatoire de leurs comptes. Le Comité estime qu'une réponse appropriée ne peut résulter que d'un faisceau d'interventions. « À l'évidence, l'entreprise qui, en l'absence d'obligation de commissariat aux comptes, aurait opté pour un " audit légal PE " se trouverait dans un environnement où le professionnel indépendant désigné serait en mesure d'alerter le chef d'entreprise à l'occasion de l'émission de son rapport sur les risques et de son attestation spécifique sur la situation financière de l'entreprise. » On aura ainsi noté que les entreprises constituant le coeur de cible de la réforme sont précisément celles dont nous avons besoin pour dynamiser l'activité et les créations d'emplois dans notre pays. Pour une partie, il s'agit d'entreprises dont nous souhaitons le développement réel, aux côtés de nos grandes entreprises, et des entreprises de taille intermédiaire qui constituent, pour l'heure, la capacité exportatrice de notre pays. Quel

à adopter une réglementation des levées de fonds par émission de jetons, qui aident au développement d'un projet. L'achat de jetons ne vaut pas l'attribution d'actions, mais équivaut à prépayer le service lié au projet, moyennant une décote, une fois que celui-ci sera opérationnel. Nous devons encourager ces levées de fonds, mais en les entourant d'un minimum de garanties. Or, aujourd'hui, l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers est optionnel. Dans leur rapport du 12 décembre 2018 sur l'enjeu stratégique de la en France, nos collègues députés Laure de La Raudière et Jean-Michel Mis préconisent de créer un statut de tiers de confiance numérique, chargé d'assurer la protection de l'identité, des documents, des transactions et d'auditer et certifier les protocoles. Dans cet esprit, nous proposons de nommer un commissaire aux comptes habilité à délivrer un label de qualité. Son intervention sera perçue comme un gage de transparence pour les opérations de levée de fonds par émission de jetons, aussi bien par la préparation d'un document d'information fournissant de nombreuses informations financières que par la mise en place de procédures de lutte contre le blanchiment d'argent et et pour la manipulation des fonds levés. Le contenu et les modalités de l'intervention du commissaire aux comptes seront définis dans des normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice. Quel est l'avis de la commission spéciale ?

des sociétés commerciales et remplace cet audit légal obligatoire par un audit contractuel soumis au bon vouloir de la gouvernance de ces sociétés. Le présent amendement a pour objet de répondre à l'objectif de transformation de la profession de commissaires aux comptes en introduisant les contours de la nouvelle mission d'audit légal Petites entreprises et en la rendant plus attractive pour les acteurs économiques. Cet audit repose sur une analyse des risques, une prise de connaissance du système de contrôle interne et une revue analytique des états financiers et des travaux de contrôle des comptes ciblés dans les principales zones de risques.

Cet amendement vise également à donner une appellation plus positive à cet audit : plutôt que « rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion », je vous propose l'appellation « diagnostic de performance et de croissance », beaucoup plus valorisante. La parole est à M. Alain Houpert, pour présenter l'amendement

et qu'il choisit de limiter la durée de son mandat à trois ans. Nous pensons que ce dispositif sera plus clair que l'inclusion de cette disposition à l'article L. 823-3. En outre, l'amendement prévoit de nouvelles exemptions pour les missions de commissaires aux comptes mandatés pour une mission d'audit légal Petite entreprise.

L'alinéa 38 introduit des normes d'exercice professionnel déterminant les diligences que le commissaire aux comptes doit accomplir pour une mission d'audit légal Petite entreprise, qu'il exerce cette mission dans une société tête de petit groupe ou dans une filiale. Il prévoit que les normes traiteront les diligences à accomplir

reposant sur le triptyque suivant : la délivrance d'une attestation de sincérité et de régularité comptables, la remise d'un rapport prospectif sur les risques auxquels est confrontée l'entreprise et la délivrance d'attestations spécifiques à valeur ajoutée Cette mission, qui restera optionnelle pour les entreprises, vise à leur permettre de bénéficier des effets favorables attachés à l'intervention d'un professionnel indépendant et qualifié, qui est de nature à contribuer à sécuriser les tiers, mais aussi et surtout à conforter, de façon à la à la fois rétrospective et prospective, le chef d'entreprise lui-même dans ses analyses, tant en termes de gestion que de conformité et de prise en compte des risques. » Deux recommandations sont relatives au groupe : « rendre le commissariat aux comptes obligatoire pour la société faîtière d'un groupe se trouvant elle-même en deçà des seuils, dès lors que l'entité économique constituée par le groupe se situe au-delà ; soumettre les filiales de groupe à des diligences proportionnées : réalisation d'un " audit légal Petite entreprise " pour les filiales importantes du groupe, définies comme celles dont le chiffre d'affaires dépasse 4 millions d'euros, soit 50 % du nouveau seuil, diligences spécifiques fondées sur le jugement du commissaire aux comptes de la société faîtière et réalisées par lui pour les autres filiales. « À l'issue de la période transitoire de trois ans, le nouveau dispositif s'appliquerait selon les modalités exposées précédemment. Le comité considère qu'une telle mesure placerait entreprises et commissaires aux comptes sur un pied d'égalité, en éliminant les conséquences liées aux échéances des mandats en cours, par construction réparties de façon aléatoire

de loi. Ils répètent des dispositions qui figurent déjà dans le code de commerce sur la mission générale d'audit des commissaires aux comptes. Je rappelle que l'élaboration d'une norme d'exercice professionnel est prévue par le projet de loi. En outre, ces amendements tendent aussi à modifier le nom et le contenu du rapport sur les risques qui doit accompagner, dans ce dispositif d'audit simplifié, le rapport d'audit lui-même : il ne s'agirait plus d'un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société, ce qui relève du coeur de la mission d'un commissaire aux comptes, mais d'un diagnostic de performance et de croissance. L'avis est donc défavorable sur ces deux amendements

J'en demande le retrait. M. Lalande propose de supprimer les références à la mission d'audit des sociétés mères ou à la mission d'audit simplifié pour les petites entreprises. Or ces références sont nécessaires pour savoir sur quoi

donc dans la droite ligne de l'esprit dans lequel la profession a pu appréhender la réforme de ses activités, c'est-à-dire positivement, avec le souci de faire admette son activité comme une nécessité pour le développement des entreprises, non comme une sorte d'obligation soudain disparue. De ce point de vue, le projet de loi entretient d'ailleurs une certaine forme d'équivoque,

Le contrôle professionnel et disciplinaire des commissaires aux comptes appartient déjà au Haut conseil du commissariat aux comptes. Cet amendement n'a donc pas d'utilité. Avis défavorable. Quel est

S'agissant de ces entités, le texte prévoit que, dans cette hypothèse, les missions du comité sont exercées par un autre organe. Le présent amendement a pour objet d'inclure les sociétés de financement au bénéfice de ces dispositions, donc de simplifier le l'ensemble du dispositif.

d'évolutions très importantes du milieu des entreprises et du droit en matière d'économie, la formation des experts-comptables doit être améliorée, afin qu'ils puissent accompagner au mieux les entreprises en difficulté. Le manque de formation a été signalé, selon M. Antiste, à de nombreuses reprises par ces professionnels.

dans les procédures qu'elles engagent. C'est à l'image de ce qu'on attend des médecins, des architectes et de toutes les autres professions à hautes compétences intellectuelles et qui nécessitent des mises à jour permanentes.

Cet amendement découle assez naturellement du contenu de la réforme, plus ou moins écrite par l'article 9, et de la transposition de la directive. L'article L. 822-15 du code de commerce pose le principe du secret professionnel, élément essentiel de la déontologie des professionnels du chiffre, commissaires aux comptes ou experts-comptables. Ce secret professionnel n'est bien entendu pas pas opposable à l'expresse demande du président du tribunal de commerce compétent pour examiner une procédure collective, entre autres cas d'espèce : si le président en éprouve le besoin, il peut demander au commissaire aux comptes mandaté par l'entreprise concernée de lui faire part de ses observations, comme des éléments lui ayant servi à certifier les comptes. Au demeurant, le commissariat aux comptes emporte également une mission d'alerte, qui se conçoit aisément

? Cet amendement traite de la responsabilité des commissaires aux comptes et du respect de la justice, alors que l'article visé du code de commerce ne concerne que la levée du secret professionnel entre les commissaires aux comptes intervenant auprès de sociétés

dans le chapitre préliminaire les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale sur les missions que peuvent réaliser les commissaires aux comptes. Il tend aussi à préciser que les autres missions des commissaires aux comptes peuvent être réalisées en dehors de tout mandat de certification des comptes.

Cet amendement reprend l'une des préconisations du rapport de Cambourg sur l'activité des commissariats aux comptes, selon lequel : « Le statut légal et réglementaire du commissaire aux comptes lui confère une crédibilité élevée. Le comité rappelle en particulier les points suivants. « aux comptes est garantie par le niveau de formation requis pour son inscription initiale en cette qualité et pour la poursuite de son droit d'exercer. Sa probité et vérifiée lors de son inscription et encadrée pendant sa vie professionnelle. Son indépendance est encadrée par un code de déontologie rigoureux, garantissant qu'il ne peut se trouver, à l'égard des entités auprès desquelles il intervient, ni en situation de conflit d'intérêts, ni en auto-révision, ni en position de décideur ou de co-décideur. L'exercice de la plupart de ses missions, notamment celles qui apparentent son action à un service public, est régi par des normes d'exercice professionnel adoptées dans des conditions garantissant la prise en compte de l'intérêt général et le plus haut niveau de qualité international. Enfin, son exercice professionnel est suivi dans le cadre d'un contrôle de qualité structuré et approfondi, placé sous l'égide d'une autorité publique indépendante. « Sur ces bases, le commissaire aux comptes est le tiers de confiance par excellence dans les matières de sa compétence. S'il faut caractériser son rôle par rapport à celui de l'expert-comptable, qui est également souvent qualifié de tiers de confiance, l'on peut indiquer qu'il est tiers de confiance indépendant. C'est en effet son indépendance qui attache une valeur particulière à ses interventions et une véritable portée à ses conclusions et rapports. C'est elle qui différencie ses interventions de celles de l'expert-comptable qui opère le plus souvent en assistance et en conseil auprès de ses entreprises clientes.

et de contentieux au titre de la profession de commissaire aux comptes. Actuellement, le rapporteur général du Haut conseil et ses services ne peuvent, dans le cadre d'une enquête, obtenir de documents ou d'informations que si les pièces sont relatives à la mission de certification des comptes, ou à toute prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes et entités dont il certifie les comptes. Pourtant, les pouvoirs de sanction du Haut conseil portent également sur les manquements à l'honneur et à la probité. probité. Autrement dit, les pièces qui permettent de démontrer l'existence de ces manquements ne sont pas nécessairement en lien avec une mission de certification de comptes en particulier. Telle est la limite que le présent amendement vise à modifier.

n° 766 vise à mieux coordonner le regroupement des commissions régionales de commissaires aux comptes. Actuellement, ce regroupement a lieu sur l'initiative de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Nous proposons que l'initiative appartienne au garde des sceaux

les fonctions et la place du Haut conseil. Un premier délai permettrait au garde des sceaux de demander au Haut conseil de rédiger le projet de norme, dans le cas où la commission mixte n'y serait pas parvenue. Un second délai permettrait au Haut conseil

être menée à bien en 2019. Cet amendement vise à accompagner cette réorganisation et à éviter la liquidation des compagnies régionales dissoutes, ainsi que les montages juridiques complexes, pour les compagnies absorbantes.

En vertu de l'article 9 du présent texte, les sociétés d'économie mixte locales qui ont le statut de société anonyme ne se verraient plus imposer la désignation d'un commissaire aux comptes si elles se trouvent en deçà des nouveaux seuils. Or ces sociétés gèrent des fonds publics pour des montants très significatifs. Dès lors, il convient de prendre en compte cette spécificité et de conserver pour ces SEM, en toute hypothèse, l'obligation de désigner un commissaire aux comptes.

Ces dispositions découlent, si l'on peut dire, du développement des formes de financement participatif dans notre pays. Il s'agit tout simplement d'étendre les compétences des commissaires aux comptes,

Il s'agit, selon nous, d'un sujet d'une importance majeure pour nos concitoyennes et nos concitoyens : c'est celui de la juste qualification et donc de la juste protection du travail. du travail. Nombre d'entre vous auraient d'ailleurs approuvé notre objectif : redonner à l'entrepreneuriat ses lettres de noblesse ! Ne nous méprenons pas. Il n'est pas question ici d'embrasser une doctrine encourageant la sortie du salariat, mais, au contraire, d'en clarifier les contours. toute fuite du statut de salarié vers une indépendance purement nominale et formelle aboutit à une dégradation des conditions de l'entrepreneuriat ; elle nuit au vrai travail indépendant. Pour preuve, l'on dénonce aujourd'hui l'explosion du nombre d'auto-entrepreneurs, qui favorise la concurrence déloyale et le salariat déguisé.

conduit comme nombre de ses collègues à prendre des risques toujours plus grands pour gagner un salaire toujours plus misérable. Il est donc nécessaire de proposer une définition légale du salariat, afin de mettre un terme aux stratégies des plateformes, lesquelles sont dangereuses pour l'économie du pays et pour la vie des travailleurs. C'est pourquoi nous avions proposé, avec cet amendement, d'inscrire dans la loi ce qui est déjà acté dans les prétoires depuis l'arrêt : les travailleurs des plateformes doivent être considérés pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des salariés.

Toutefois, il est primordial de pouvoir identifier et contrôler les activités professionnelles d'un micro-entrepreneur, quel que soit le montant de son chiffre d'affaires ; et seul un compte bancaire séparé permet Au-delà du risque de dissimulation de tout ou partie de l'activité, cet article pourrait créer une forme de concurrence déloyale au détriment d'entreprises déjà installées et créatrices d'emplois. À l'heure où l'État tente de renforcer les moyens de contrôle pour prévenir les fraudes, il serait difficilement compréhensible de favoriser l'émergence d'un pan d'activité en dehors de tout contrôle. De plus, le compte bancaire séparé revêt un caractère éducatif pour les créateurs d'entreprise.

pour les micro-entrepreneurs.

« Il faut éviter qu'un entrepreneur se heurte à la complexité administrative, à la sur-réglementation ou à toute sorte de difficultés, lorsqu'il veut créer une activité dans une cité ou sur internet. Cela vaut pour tous les créateurs d'entreprise, qu'il s'agisse de retraités ou de salariés, qui souhaitent développer une activité en dehors de leur travail. C'est à leur profit que nous voulons instituer le régime de l'auto-entrepreneur dans notre pays. Ce régime présente le grand avantage de rendre les choses plus simples. » Mes chers collègues, en ce sens, nous vous proposons

pas les mêmes charges que son employeur. Cela peut donner lieu à une concurrence déloyale, notamment en ce qui concerne la fixation du prix des prestations. Un artisan doit en effet fixer un prix lui permettant d'être assuré, de couvrir ses frais salariaux, d'assumer ses responsabilités envers ses clients en termes d'assurance et de lui procurer un revenu. Un micro-entrepreneur, également salarié, n'est pas soumis à l'ensemble de ces contraintes, son revenu étant déjà assuré par son activité salariée. Au sein du même secteur économique, cette distorsion de concurrence peut également emporter des conséquences sur la pérennité des petites entreprises, voire sur les emplois. En outre, si la loi oblige le micro-entrepreneur à demander l'autorisation du chef d'entreprise pour exercer une activité couplée, force est de constater que cette règle n'est pas souvent respectée.

De plus, je rappelle qu'un salarié qui souhaiterait mener une activité indépendante dans le même secteur que son employeur doit en demander l'autorisation à ce dernier. S'il ne le fait pas, il peut être poursuivi. Sur le second point, la limitation du statut de micro-entrepreneur à deux ans pourrait avoir pour conséquence de priver d'activité des micro-entrepreneurs qui ne pourraient pas trouver d'emploi ou mener une activité artisanale

le scepticisme. Je lui rends hommage, parce que j'estime que cela a permis une libération des capacités de beaucoup de Français qui voulaient travailler de manière plus autonome. en partie à la question de M. Gay sur le salariat. La réalité, c'est que des millions de nos compatriotes veulent travailler davantage pour bénéficier d'une meilleure rémunération à la fin du mois

pourtant un service public réparti sur l'ensemble du territoire national dans un souci d'égalité de tous nos concitoyens. Comme vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, les chambres consulaires existent depuis le XVI siècle, elles font partie de notre culture et sont véritablement utiles en matière de formation comme de conseil aux entreprises. Vous nous dites qu'elles doivent se réinventer, mais c'est leur asphyxie que vous organisez aujourd'hui. En effet, vous ne cessez de réduire leurs moyens près de 400 millions d'euros de ressources publiques en moins d'ici à 2022, une baisse qui entraînera la suppression de près de 2 500 équivalents temps plein, mais aussi la régionalisation des chambres de commerce Pourtant, c'est une politique d'accompagnement fine de l'ensemble du territoire qu'il faudrait privilégier. Comme le rappelait justement André Chassaigne à l'Assemblée nationale, dans nos territoires ruraux ou dans les petits bassins industriels, les CCI constituaient constituaient un véritable levier de développement économique en raison de leurs liens avec la société civile et les élus. Elles avaient un rôle de proximité déterminant. Or aujourd'hui, de réforme en réforme, coupe budgétaire après coupe budgétaire, elles n'ont plus les moyens de remplir cette fonction pourtant indispensable pour un territoire, mais aussi, et surtout, pour les petites et moyennes entreprises. Outil d'accompagnement des entreprises, de leur installation, de la formation de leurs personnels, de leur expansion, elles seront finalement transformées en simple guichet. Les PME perdent ainsi petit à petit, décennie après décennie, des accompagnateurs déterminants pour leur activité. Ne nous y trompons pas, avec les dispositions des articles 13 et suivants, les chambres de commerce et d'industrie de certains territoires vont disparaître. À force de prôner une répartition équilibrée des acteurs économiques sur nos territoires parla mutualisation des moyens et de penser que l'échelon régional, toujours plus éloigné, est le plus pertinent pour organiser cette mutualisation, vous dépouillez les territoires les plus fragiles et vous en faites des territoires abandonnés de la République. Cela n'est pas acceptable.

la libéralisation introduite par le recours à un personnel de droit privé et la redéfinition de la mission des CCI dans une optique concurrentielle. Nous pensons tout d'abord que le type d'accompagnement économique assuré par les CCI exige du personnel présent dans la durée. Or le statut de droit public garantit précisément la présence au sein des structures d'un personnel pérenne, qui connaît le territoire, ses chefs d'entreprise, ses leviers de développement. Voilà pourquoi il s'agit bien d'efficacité. Ensuite, loin de rationaliser le réseau consulaire au service des entreprises de l'ensemble de notre territoire dans ses différentes réalités, cet article se limite à gérer la pénurie des ressources allouées à ce réseau

les ressources fiscales ont baissé de plus de 40 % depuis 2013. Il s'agit donc d'inciter les CCI à se financer elles-mêmes en vendant des produits sur des marchés concurrentiels. Cela ne correspond pas à notre vision d'un véritable accompagnement des PME. La

On peut citer, notamment, les mesures qui visent au développement de l'activité des CCI dans le champ concurrentiel et l'obligation de recrutement de salariés de droit privé. Cette réforme est guidée par le désengagement de l'État et l'urgente nécessité de trouver d'autres moyens pour faire vivre les CCI,

Pour ces CCI rurales, la taxe affectée représente une part très importante des ressources : jusqu'à 65 %. Il leur sera donc très difficile de basculer vers un financement par prestations. Sans un système de péréquation efficace, ces CCI risquent à terme de disparaître. Le projet de loi ne prend pas suffisamment en compte les besoins des très petites entreprises, les TPE, sur les territoires fragiles, aussi bien dans le rural que dans les quartiers de la politique de la ville. Cette réforme se fait donc avant tout au détriment des CCI rurales dont l'existence même se trouve menacée à très court terme, ce qui est un très mauvais signal au regard des événements des

tout ce qui fait des départements des territoires vivants, animés et qui peuvent rendre des services attendus tant par les particuliers que par les entreprises. Je vous invite à changer d'orientation et à vous tourner vers une autre politique, plus départementalisée.

Monsieur le ministre,

la disparition des CCI. Je maintiens chacun des mots que j'ai prononcés, qu'ils plaisent ou non : j'ai voulu mettre un terme à cette manière de traiter les chambres consulaires qui appartiennent depuis plusieurs siècles à notre histoire économique et auxquelles je suis attaché.

nous avons préféré construire d'autres modalités de financement, notamment par des prestations financées. Je rends un hommage appuyé à tous les présidents de CCI que j'ai reçus à plusieurs reprises, soit en assemblée générale,

la possibilité d'affiliation de tous les salariés des CCI au régime général d'assurance chômage. Selon moi, c'est la clé du succès de cette transformation.

parce que le président de la CCI de Rennes vous a écrit il y a un mois et m'a confié un double de la lettre. Vous n'avez pas répondu, c'est normal, vous n'avez pas eu le temps. Dans cette lettre, il ne vous dit pas du tout qu'il est satisfait

et dire qu'il faut que l'État assume les conséquences de ses actes. Je ne me rendrai pas complice d'une opération consistant, à terme,

je n'ai pas bien compris : « Monsieur le sénateur, vous connaissez les nombreuses activités de notre CCI au bénéfice de nos entreprises et de nos territoires. Nous avons d'ailleurs régulièrement l'occasion d'agir ensemble- merci -pour stimuler le développement économique et renforcer l'attractivité de la Marne et nous tenons à vous en remercier. » Jusqu'ici, tout va bien ! « Je dois cependant vous alerter sur la grave menace qui pèse sur les CCI, à laquelle notre établissement public départemental n'échappera pas, malgré ses nombreuses réussites. En effet, après avoir connu une perte de la moitié de nos ressources fiscales en cinq ans- là, on vous rejoint, monsieur le ministre -, le Gouvernement vient de nous annoncer que nous allons voir ces ressources une nouvelle fois divisées par deux dans les quatre ans qui viennent. Cette annonce a été faite au mépris des engagements de stabilité qui avaient été pris par le ministre Le Maire il n'y a même pas un an.

Il est absolument indispensable que cet élément de proximité perdure. Les chambres de métiers et les chambres de commerce, cela a été dit ici, ont cet avantage de savoir répondre aux besoins de leurs ressortissants et leur enlever cette possibilité

Le projet de loi PACTE va fortement modifier l'organisation du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Les CCI connaîtront une réduction importante de leurs ressources, qui pose la question d'une réelle péréquation au bénéfice des CCI territoriales implantées dans des départements ruraux. Les CCI rurales, si elles ne bénéficient pas d'un système de financement minimal spécifique, nécessaire au maintien de leurs activités d'appui et de soutien des entreprises, ne survivront pas à ces nouvelles réformes. Ce projet est un pas de plus vers un risque de régionalisation du réseau des CCI et la mort annoncée des actions de soutien adaptées aux territoires les plus fragiles. « Les CCI territoriales rurales restent encore une fois les plus fragiles et les plus dépendantes de la ressource fiscale.

la commission des lois a émis, lors de sa réunion du 29 janvier 2019, un avis favorable- 13 voix pour, 5 voix contre -à la nomination de Mme Marie-Laure Denis à la présidence de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. conformément aux mêmes dispositions, la commission de la culture a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable à la nomination de M. Roch-Olivier Maistre- 26 voix pour, aucune voix contre -à la présidence du Conseil supérieur de l'audiovisuel.